Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question porte sur les entreprises adaptées et leur situation financière. L'entreprise adaptée est une entreprise à but social, composée majoritairement de travailleurs handicapés, mais dont le statut- les droits et les devoirs -ne diffère pas L'entreprise adaptée, intervenant sur un marché concurrentiel, est soumise aux mêmes contraintes de rentabilité et d'efficacité économique que toute autre entreprise. Mon département, le Pas-de-Calais, compte 13 entreprises

Si cette volonté est tout à fait honorable, madame la ministre, elle ne correspond pas aux réalités de terrain : aujourd'hui, dans mon département, les entreprises adaptées emploient la plupart du temps des personnes atteintes de déficience cognitive et qui ont d'énormes difficultés à trouver un emploi en milieu ordinaire. La diminution des aides, de l'ordre de 10 millions d'euros par an, accroîtra les difficultés sociales déjà importantes sur mon territoire, et ce d'autant que, selon certaines études, le retour à l'emploi permet un gain social égal à 11 000 euros par travailleur handicapé par rapport à une situation de non-emploi. Je souhaite également préciser que l'État intervient financièrement pour compenser, et non assister les entreprises adaptées. En effet, chaque euro investi par l'État est récupéré par le biais des cotisations et des impôts publics engendrés par le retour à l'emploi. Vous comprendrez, madame la ministre, que les dernières mesures prises par le Gouvernement inquiètent fortement le secteur des entreprises adaptées. Je souhaiterais donc vous interpeller sur trois points. Premièrement, si l'on peut se féliciter du report de la réforme au 1 janvier 2019, comptez-vous engager, à la rentrée de septembre, un véritable processus de concertation

Troisièmement, l'État souhaite que les entreprises adaptées s'orientent davantage vers l'insertion. Comptez-vous donc prendre en compte dans les prochains contrats d'objectifs triennaux la particularité des handicaps intellectuels et psychiques et intégrer des modalités spécifiques d'accompagnement des entreprises adaptées concernées ? La parole

Corbisez, les entreprises adaptées jouent un rôle essentiel dans la stratégie d'inclusion dans le travail et dans l'emploi, qui est un facteur d'émancipation pour tous.

Je suis donc convaincue de la place fondamentale des entreprises adaptées dans notre stratégie globale d'émancipation par le travail et d'inclusion par l'emploi. C'est pourquoi j'ai procédé, pour l'année en cours, à une hausse du budget des aides au poste pour les entreprises adaptées

probablement intégrer d'autres structures. Cette concertation est construite autour de deux axes. Le premier axe consiste à réaffirmer la vocation économique et sociale des entreprises adaptées, vous l'avez soulignée. Il s'agit de valoriser leur « savoir-faire inclusif », construit autour du triptyque : « situation d'emploi réelle, formation, accompagnement personnalisé ». Le second axe consiste à innover en expérimentant de nouvelles approches du parcours professionnel des travailleurs handicapés,

C'est une transformation ambitieuse et partagée que nous allons mener et qui marquera, je l'espère, le point de départ d'un développement inégalé de l'emploi des personnes handicapées. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour répondre à Mme la ministre.

Le tribunal a refusé d'homologuer ce prénom, s'appuyant sur une circulaire de la garde des sceaux du 23 juillet 2014 relative à l'état civil, qui régirait l'usage des signes diacritiques et des ligatures dans la langue française.

qui a trait à la reconnaissance du « tilde » dans les actes d'état civil. Le principe de liberté de choix du prénom d'un enfant, effectivement consacré par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et au droit de l'enfant

dont le Conseil constitutionnel a déduit que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage.

si ce signe a été refusé par le tribunal de grande instance de Quimper en septembre dernier, les parents de l'enfant ont fait appel du jugement et la cour d'appel de Rennes n'a pas encore rendu son arrêt. Mais je tiens à préciser que les textes en vigueur, confortés par la jurisprudence, n'excluent pas que les communes puissent délivrer des livrets de famille bilingues, dès lors que les livrets de famille sont rédigés en langue française, dans le respect des règles précédemment évoquées, et que la traduction en langue régionale fait simplement office d'usage.

sapeurs-pompiers professionnels ou personnels administratifs techniques et spécialisés, correspondant à 0,9 % de leur masse salariale, ainsi qu'une sur-cotisation affectée spécifiquement à la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, correspondant actuellement à 0,86 % de la masse salariale des sapeurs-pompiers professionnels. La formation des officiers sapeurs-pompiers étant exclusivement assurée par l'établissement national de formation des sapeurs-pompiers, cette sur-cotisation est intégralement

Aussi, je souhaiterais savoir, madame la ministre, si le Gouvernement envisage de faire de l'ENSOSP l'organisme collecteur unique des cotisations des SDIS pour le financement des actions de formation destinées aux sapeurs-pompiers,

sur le financement des collectivités locales, est dirigé vers le CNFPT. Compte tenu de leur spécificité, les formations opérationnelles pour les officiers

en tant que financeur. À ce titre, le Centre verse à l'ENSOSP une part de la cotisation précitée, ainsi qu'une sur-cotisation spécifique provenant des SDIS pour le financement des formations des officiers.

attentifs aux interrogations soulevées, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et le président de l'Association des maires de France, l'AMF, ont demandé au président du CNFPT de leur apporter tous les éléments utiles pour la compréhension de l'utilisation des fonds récoltés, soit une transparence totale. Dans le même temps, le CNFPT s'est engagé à assurer sur ses fonds propres le versement des sommes correspondant au montant de la sur-cotisation et à la scolarité de la première promotion d'élèves-colonels en 2018. Dans ce contexte, le Gouvernement n'entend pas prendre l'initiative d'une modification structurelle d'un dispositif reposant sur la capacité de concertation des acteurs. En tout En tout état de cause, le ministère de l'intérieur reste extrêmement attentif à la pérennité de financements adaptés à la mise en oeuvre des formations de haut de niveau qui sont la marque de l'excellence du système français de sécurité civile. La parole est à M.

rejeter en bloc cette mesure. En revanche, j'ai défendu l'idée- et j'avais écrit un courrier au Premier ministre dans ce sens -de conserver sur quelques axes structurants une vitesse de 90 kilomètres

porte sur la protection sociale des agents territoriaux sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. L'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 prévoit en effet une prise en charge en cas d'accident des sapeurs-pompiers volontaires, qu'ils soient fonctionnaires, titulaires, stagiaires ou même militaires, non pas par le service départemental d'incendie et de secours, ou SDIS, mais par la collectivité territoriale dont ils dépendent. Ils bénéficient alors du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. Ces frais, souvent importants, doivent alors être supportés par les communes, qui se retrouvent à payer pour un accident sans aucun rapport avec le service rendu par ces personnes en tant qu'agents communaux.

En octobre 2013, le ministre de l'intérieur avait signé un plan d'action pour les sapeurs-pompiers volontaires, qui prévoyait, dans sa mesure n° 6, la généralisation, par le biais d'une modification de la loi de 1991, de la prise en charge de la protection sociale par les SDIS. Cette volonté affichée ne s'est pas traduite à ce jour par une modification de la loi. Si l'article 19 de la loi de 1991 était maintenu en l'état, le statut de sapeur-pompier volontaire pourrait représenter un réel frein à l'embauche dans les collectivités territoriales. Notre collègue Catherine Troendlé, dont je tiens ici à souligner l'excellent travail, vous a remis le 23 mai dernier son rapport sur la mission volontariat, elle préconise- c'est la proposition 18 -de généraliser la prise en charge par les SDIS de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires employés dans la fonction publique en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Aussi, madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer si le Gouvernement entend donner une suite favorable à ces préconisations afin de sécuriser financièrement les collectivités territoriales qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires ?

Déjà touchée à deux reprises au cours des trois derniers mois, la commune de Bressols a récemment fait l'objet d'un vol, pour un préjudice de 14 000 euros. De ce fait, les entreprises locales de Tarn-et-Garonne pâtissent de cette situation. jours ont été nécessaires pour établir la connexion téléphonique et internet à la suite de ce vol dans la commune de Bressols. Cela a privé 3 700 habitants et quelque cinquante entreprises situées sur les quatre zones d'activité de cette commune de tout moyen de communication.

sénateur, les vols de métaux en France font l'objet de la plus grande attention de la part du Gouvernement. Le phénomène présente en effet une sensibilité toute particulière, au regard du double préjudice subi par les entreprises et par les particuliers. Le premier préjudice est lié à la valeur des métaux dérobés. Cela constitue une perte pour l'entreprise ou la collectivité. Leur nécessaire remplacement est donc un coût pour la victime. Le second préjudice, plus important encore, correspond aux conséquences induites par ces vols, notamment celles liées à la communication ou à l'alimentation électrique, comme vous venez de le rappeler. Force est de constater que ces vols de métaux sont le fait non pas d'individus isolés, mais de réseaux criminels organisés, notamment originaires de l'Europe de l'Est. Face à cette problématique, le ministère de l'intérieur possède une stratégie de longue date. Ainsi, dès la fin de l'année 2006, la gendarmerie nationale a mis en place un plan d'action destiné à lutter contre les vols de métaux. Un rôle de coordination a été confié à l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, l'OCLDI. Sur le plan opérationnel, le ministère de l'intérieur met ainsi en place une approche globale fondée, d'une part, sur la prévention des phénomènes et le partenariat avec les entreprises privées, et, d'autre part, sur le démantèlement des groupes criminels organisés. Dans ce contexte, de nombreux partenariats sont mis en place avec les sociétés victimes de vols de métaux. Six conventions régionales ainsi ont été élaborées entre la société Orange et les régions de gendarmerie de Midi-Pyrénées, de Bretagne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Lorraine, d'Aquitaine et, récemment, d'Île-de-France. Par ailleurs, une action volontaire est menée permettant de démanteler ces groupes criminels organisés itinérants, ce qui signifie interpeller les auteurs, mais également les receleurs et éventuellement les donneurs d'ordre. Très récemment, à la fin de 2017, l'OCLDI a ainsi procédé sur la région toulousaine à l'interpellation de onze individus majoritairement originaires de Roumanie. Ces malfaiteurs, tous écroués, sont impliqués dans cent cinq faits de vol commis au sein des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, avec l'installation d'élingues pour dérober les câbles de la société Orange. Enfin, le problème n'est pas

Ainsi, sur la base de ces dispositions, des syndicats d'énergie détenteurs de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité se sont vu confier par leurs collectivités membres des prérogatives liées à la maîtrise d'ouvrage des installations d'éclairage public. ENERGIE Eure-et-Loir assure désormais la gestion quotidienne de plus de 32 000 foyers lumineux pour le compte de 165 communes. Au cours des dernières années, ce syndicat a massivement investi sur les réseaux d'éclairage public, pour remplacer les installations vétustes et très consommatrices d'électricité, en proposant des solutions peu énergivores et innovantes. Pour procéder à ces investissements, le syndicat d'énergie a eu recours au mécanisme de fonds de concours appelés auprès de ses communes membres. Or il semblerait que la Direction générale des collectivités locales, ou DGCL, remette en cause le régime de ces fonds de concours s'agissant des syndicats d'énergie. Si cette position venait à être confirmée, elle serait de nature à ruiner les efforts déployés localement. Monsieur le secrétaire d'État, j'aimerais savoir pour quelles raisons et sur quel fondement juridique la DGCL restreint l'utilisation du mécanisme des fonds de concours par les syndicats d'énergie et leurs collectivités adhérentes, dès lors que ces établissements publics de coopération interviennent

la position du Gouvernement sur l'utilisation du mécanisme des fonds de concours par les syndicats d'énergie. Le rôle des groupements de communes est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres, la commune et le groupement ne pouvant pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est l'une des conditions nécessaires à la clarté de notre organisation locale. C'est sur ce principe que je m'appuie pour vous répondre. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. de coopération intercommunale, ou EPCI, à fiscalité propre. Pour les autres groupements, comme les syndicats de communes, ils ne sont autorisés que dans des cas très particuliers. Il peut ainsi être fait usage des fonds de concours pour trois autres compétences prévues de manière dérogatoire dans le code général des collectivités territoriales : par un syndicat mixte ouvert pour la gestion et la construction des ports autonomes ; par un syndicat intercommunal pour la distribution publique d'électricité ; par un syndicat mixte ouvert pour l'établissement des réseaux publics de communication électronique. Le législateur a établi des critères organiques et fonctionnels très clairs pour encadrer l'usage des fonds de concours. Dans le cas que vous citez des syndicats intercommunaux compétents en matière d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, ceux-ci peuvent, afin de financer la réalisation ou d'assurer le fonctionnement d'un équipement public local, percevoir ou verser à leurs membres des fonds de concours. Le renvoi opéré par l'article L. 5212-26 à l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales restreint cependant le champ d'action du fonds de concours à la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité du syndicat. Les autres compétences exercées sont donc exclues. Le texte est très clair, et doit être d'interprétation stricte, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État en la matière. Dans ce cas ... La compétence d'autorité organisatrice du réseau de distribution d'électricité étant une compétence spécifique, distincte par exemple de celle en matière d'éclairage public, les travaux réalisés en matière d'éclairage public ne peuvent en effet être financés par le biais des fonds de concours. Cela ne signifie cependant aucunement que ce type de travaux ne peut être financé.

Le cuivre est l'un des seuls produits minéraux autorisés par la réglementation européenne pour lutter contre les bactéries et autres maladies fongiques. Il est utilisé aussi bien en viticulture biologique qu'en viticulture dite « conventionnelle », mais également pour les cultures maraîchères et même fruitières. Concernant la viticulture biologique, un rapport de l'Institut national de la recherche agronomique, ou INRA, publié en janvier 2018, montre que, à court terme le remplacement du cuivre n'est envisageable, la piste génétique restant une stratégie à moyen terme. Ainsi, à ce jour, seule une gestion optimisée des doses en fonction des circonstances de l'année permettrait de diminuer l'impact du cuivre tout en lui conservant son efficacité. Il faudra probablement attendre quelques années avant que des solutions de biocontrôle ou que des variétés résistantes ne puissent remplacer le cuivre. Sans cuivre, ou en quantité insuffisante, les producteurs ne pourraient que se détourner du mode de production biologique, ce qui serait contradictoire avec les objectifs fixés par les pouvoirs publics. Concernant la viticulture conventionnelle, la consommation de cuivre devrait mécaniquement continuer à augmenter compte tenu de l'orientation souhaitée vers une forte réduction des produits classés « substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction Le 16 janvier 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou EFSA, a transmis à la Commission européenne ses conclusions en vue d'une nouvelle homologation. Celle-ci devra se prononcer avant le 31 janvier 2019 sur une nouvelle approbation du cuivre au niveau au niveau européen comme substance active dans la protection des plantes. Sans renouvellement de l'autorisation d'utilisation du cuivre, la filière viticole française se trouverait dans une impasse technique, avec des incidences importantes pour la filière biologique viticole. par hectare et par an lissée sur cinq ans, soit 0,6 gramme par mètre carré, est la seule qui soit soutenue par la profession. L'élément de lissage est très important, car il permet de faire face à une pression des maladies, qui change d'année en année en fonction des aléas climatiques. Enfin, pour la profession, il serait inconcevable d'interdire immédiatement l'usage du cuivre, utilisé depuis plus d'un siècle et demi, sans solution de rechange efficace et à un coût acceptable. Monsieur le ministre, pouvez-vous me préciser quelle position compte prendre la France à l'échelon européen concernant le renouvellement de l'homologation du cuivre ?

Vous me demandez quelle sera la position du Gouvernement concernant le renouvellement de l'approbation européenne du cuivre, en tant que produit phytopharmaceutique. Le cuivre et ses différents composés, comme la bouillie bordelaise, sont connus de longue date comme produits de protection des plantes, en particulier pour traiter le mildiou de la vigne ou de la tomate. vous le savez comme moi, le cuivre est persistant dans l'environnement et toxique, ce qui le classe dans la catégorie des substances dont on doit envisager la substitution chaque fois que c'est possible. L'approbation européenne expire en janvier 2019. L'évaluation scientifique de l'EFSA conclut que certaines données sont manquantes et que des risques sont identifiés pour les utilisations demandées à 6 kilogrammes par hectare et par an sur la vigne et les tomates notamment. Cependant, elle indique qu'il est possible de limiter les risques, en réduisant les doses utilisées. Le Gouvernement est favorable au renouvellement de l'approbation du cuivre. Il sera toutefois nécessaire

dans le cas des cultures pérennes comme la vigne. Il s'agit d'autoriser un dépassement limité de la quantité admise au cours d'une année, à condition que l'apport total sur l'ensemble de la période ne dépasse pas la quantité maximale permise. Si elle est retenue, cette possibilité de lissage nécessitera toutefois,

les différentes filières de l'agriculture conventionnelle et surtout de l'agriculture biologique, il est nécessaire d'accélérer les travaux pour réduire son utilisation en protection des cultures. L'expertise scientifique collective de l'INRA publiée en en janvier 2018 a identifié des leviers d'action qui permettraient de réduire les quantités utilisées, sans remettre en cause l'efficacité de la protection phytosanitaire. Les différentes combinaisons de moyens, y compris la « reconception » des systèmes de culture- assolement ; choix de variété ; conditions de semis -doivent désormais être validées avant d'être généralisées.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Vous avez compris l'importance du cuivre pour toutes ces productions.

Pour ce faire, selon l'article 79 du règlement européen 1107/2009, la Commission européenne doit tout d'abord recueillir l'avis des États membres, représentés au comité permanent européen de la chaîne alimentaire et de la santé animale. À ce jour, la France, interrogée, ne s'est toujours pas positionnée sur cette question. Aussi, monsieur le ministre, il faut nous dire aujourd'hui, dans cet hémicycle, quelle réponse le Gouvernement compte apporter à la filière viticole dans la prolongation de l'homologation du cuivre agricole. Quelle réponse sera indiquée à à l'Europe ? Le constat est simple : il n'existe à ce jour aucun autre substitut crédible permettant l'abandon du cuivre en agriculture. Ce fongicide reste l'unique solution de substitution aux produits CMR pour les exploitations viticoles traditionnelles. Plus encore, en viticulture biologique, le cuivre est l'un des seuls produits minéraux homologués pour lutter contre le mildiou, maladie de la vigne pouvant entraîner des pertes de récoltes considérables si elle n'est pas combattue. À terme, la filière viticole s'est engagée à se défaire du cuivre. Les exploitants adoptent un usage raisonné et éclairé de cette fameuse « bouillie bordelaise » et soutiennent activement les recherches conduites pour développer des alternatives de biocontrôle ou de cépages plus résistants. L'utilisation du cuivre est donc en constante diminution, mais les exploitants viticoles ont encore besoin d'un peu de temps pour s'en affranchir. Un temps d'autant plus précieux pour la profession que la succession d'épisodes pluvieux a considérablement augmenté le risque de propagation du mildiou ces dernières années, dans plusieurs de nos terroirs. Pour les exploitations viticoles biologiques, la limitation actuelle à 6 kilogrammes de cuivre par hectare et par an, lissée sur cinq ans, semble offrir aux opérateurs un compromis de protection acceptable. C'est donc le cadre que vous devez préserver Aussi, monsieur le ministre, la France portera-t-elle la voix de ses viticulteurs auprès de la Commission européenne ? Prônerez-vous le maintien des conditions actuelles d'utilisation du cuivre agricole ? La

Le Gouvernement, je le répète, est favorable au renouvellement de l'approbation du cuivre. Il sera toutefois nécessaire de réduire les quantités utilisées pour maintenir le risque à un niveau acceptable.

précédente, illustrent la volonté du Gouvernement d'accompagner la filière, de construire une trajectoire, de ne pas mettre les producteurs au pied du mur et d'essayer de faire en sorte

Cela va tout simplement condamner la viticulture biologique, à Bordeaux et ailleurs, les années de pluie et au-delà. Au moment même où vous axez votre politique sur les certifications environnementales et le bio, ce que nous ressentons comme un acte très positif, vous condamnez cette même agriculture biologique par une décision ambiguë sur le cuivre. C'est une ligne politique incompréhensible. Les viticulteurs sont des chefs d'entreprise responsables. Ils n'ont aucune volonté d'empoisonner les gens ou la terre, mais ils doivent trouver le meilleur compromis entre la qualité du produit et les conditions de sa production. Nous vous demandons donc d'autoriser une utilisation du cuivre de 30 kilogrammes sur cinq ans lissés. Ainsi,

Nous progressons dans la recherche contre le mildiou, mais, vous le savez, nous n'avons pas encore la solution miracle pour remplacer le cuivre. Aussi, prenez une décision responsable, permettez aux viticulteurs d'assurer leurs productions dans des conditions décentes de protection de la vigne, de la terre

personnes handicapées. Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, ma question porte sur les délais de renouvellement des cartes de stationnement pour personnes en situation de handicap. Depuis le 1 janvier 2017, les cartes de stationnement pour handicapés sont progressivement remplacées par la carte mobilité inclusion, hormis en ce qui concerne les invalides de guerre. Les cartes mobilité inclusion, qui sont plus sécurisées, sont imprimées directement par l'Imprimerie nationale et non plus au niveau des maisons départementales des personnes handicapées. Ainsi, les délais actuels sont passés à six mois en moyenne, après constitution d'un dossier complet. De nombreuses personnes en situation de handicap sont temporairement privées de leur droit à stationner sur les places handicapées. Le fait d'apposer une carte dont la date de validité est dépassée depuis moins de six mois n'offre aucune garantie, en l'absence de directive officielle. Le risque est accru dans les villes où les infractions au stationnement sont verbalisées par des employés de sociétés privées

carte de priorité et la carte de stationnement pour personnes handicapées. Nous avançons. Je rappellerai, en préambule, que la mise en place d'une carte unique en substitution de trois cartes préexistantes constitue une vraie simplification

En outre, la carte mobilité inclusion est dorénavant fabriquée et personnalisée par l'Imprimerie nationale, qui dispose d'une grande expérience en matière de fabrication de titres sécurisés et met en oeuvre des processus de production modernisés et automatisés. Le transfert de la production de ces cartes à l'Imprimerie nationale concourt ainsi à la sécurisation des titres et à la lutte contre la fraude à la carte de stationnement, dont les premières victimes sont les personnes handicapées. Je veux vous rassurer sur les délais de délivrance de la CMI, qui ne correspondent pas à ceux qui sont issus du suivi régulier effectué par les services du ministère et en particulier par la Direction générale de la cohésion sociale, en lien avec l'Imprimerie nationale. À compter de la réception de la photo du bénéficiaire par l'Imprimerie nationale, donc lorsque le dossier est complet pour permettre la personnalisation de la carte, le délai moyen d'expédition des CMI est, sur les cinq premiers mois de l'année, de 4,58 jours exactement. Ces délais sont donc sans rapport avec le délai de six mois que vous évoquez. de six mois que vous évoquez. Par ailleurs, le délai d'envoi du courrier d'appel photo, c'est-à-dire le délai entre la réception de la commande de la carte et l'envoi du courrier par lequel l'Imprimerie nationale demande au futur bénéficiaire sa photo, est de moins d'un jour.

Monsieur le secrétaire d'État, à l'origine de ma question, il y a les fins de non-recevoir récurrentes du consulat de France à Casablanca aux demandes de visa de Mme Gracia Fuamba, demeurant régulièrement au Maroc, visas qui lui sont nécessaires pour rejoindre en France son compagnon, français et père de l'enfant qui vit actuellement avec elle. Constatant que ces demandes ont été instruites par une société privée pour le compte du consulat général, qu'il n'a été opposé auxdites demandes aucune raison sérieuse, constatant l'impossibilité de joindre cette entreprise et l'impossibilité d'obtenir des réponses autres que routinières de notre consul général à Casablanca, je me suis résolu à vous poser en direct les deux questions deux questions suivantes : qu'est-ce qui s'oppose à la venue de Mme Fuamba en France avec son enfant ? Est-il d'usage, au Quai d'Orsay, qu'un haut fonctionnaire se moque aussi ouvertement d'un élu de la République ?

à des opérateurs privés. Certes, des prestataires extérieurs sont chargés de prendre des rendez-vous et de collecter un certain nombre de pièces pour instruire les demandes.

Monsieur le secrétaire d'État, je n'aurais pas posé la question de cette façon si je n'avais pas fait l'objet d'une demande des services, pour que je fasse savoir de qui il s'agissait. J'avais donc l'espoir

Je veux simplement attirer votre attention sur un point : les motifs de refus qui m'ont été opposés sont parfaitement faux, voire ridicules, comme celui selon lequel l'enfant de deux ans n'aurait pas manifesté clairement son souhait de venir en France avec sa mère.

Monsieur le président, madame la ministre, je voudrais attirer votre attention sur la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'utilisation des eaux provenant d'une source ou d'un captage réalisé en sous-sol, par les établissements de montagne accueillant des touristes. Appréhendé sous ses angles économiques et sociaux, l'essor touristique a un impact fort en termes de développement. En s'incorporant au sein d'activités telles que l'artisanat et l'agriculture, le tourisme de montagne favorise en effet l'économie locale. Conformément aux dispositions du code de la santé publique, les établissements qui accueillent des touristes doivent respecter des principes en matière de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Toutefois, s'agissant spécifiquement des sites touristiques de montagne où les propriétaires d'auberges ou de gîtes utilisent l'eau prélevée dans le milieu naturel, il est constaté que l'application de la réglementation en vigueur varie d'un département à l'autre, ce qui ne va pas sans poser des difficultés à certains d'entre eux dans l'exercice de leur activité. Dans ce contexte, je souhaiterais connaître la doctrine en la matière et les cas dérogatoires possibles. La parole

Vous l'avez rappelé, ces structures contribuent à l'essor touristique et économique des territoires de montagne que nos concitoyens, comme les visiteurs, redécouvrent, à juste titre, L'article L.1321-1 du code de la santé publique dispose : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. Dans la mesure où les auberges et les gîtes de montagne sont des établissements recevant du public, ils sont soumis à la réglementation générale précitée. Dans certains cas, ils peuvent ne pas être raccordés au réseau public de distribution d'eau potable et utiliser leur ressource en eau privée, sous réserve de plusieurs conditions : ils doivent tout d'abord disposer d'une autorisation préfectorale, puis respecter les exigences de qualité et se soumettre au contrôle sanitaire assuré par les agences régionales de santé. Les seules exemptions à ces dispositions concernent l'utilisation d'eau en vue de la consommation à l'usage d'une famille et ne concernent en aucun cas les activités touristiques. L'application de ces règles n'a pas vocation à varier d'un département à l'autre. Aussi, à la suite de votre sollicitation, les agences régionales de santé seront alertées sur ces disparités que vous indiquez. La parole

recherche et de l'innovation. Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, j'attire votre attention sur le mode de recrutement actuel des professeurs et des directeurs de recherche dans le domaine de l'économie. Actuellement, le mode de recrutement marginalise les économistes qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la pensée économique dominante, encore dite « orthodoxe » ou. Il y a là un sujet d'importance, parce que la tradition hétérodoxe française en économie est riche en diversité et a toujours participé au rayonnement international de la France. Certains de ses représentants avaient anticipé la crise financière de 2007-2008. Les deux rapports de missions rendus en 2001 et 2014 préconisent que l'enseignement soit « incarné dans les faits, les politiques, l'histoire et les débats de société » et qu'il soit « proposé aux étudiants de premier cycle une formation pluridisciplinaire, avec spécialisation progressive, et plus tournée vers la compréhension des faits et des institutions économiques Aujourd'hui, ce défaut de pluralisme se traduit aussi par une concentration des flux financiers vers les universités et les laboratoires approfondissant la pensée dominante, ce qui renforce également les inégalités territoriales. Pour toutes ces raisons, de nombreux universitaires, notamment au sein de l'Association française d'économie politique, l'AFEP, proposent la création d'une nouvelle section, qui serait intitulée « économie, société et territoire », du Conseil national des universités, afin de valoriser les perspectives pluridisciplinaires et institutionnalistes dans l'enseignement de l'économie. Ces économistes proposent également de créer une nouvelle section, « économie et sociétés », au sein du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, pour favoriser le pluralisme et la pluridisciplinarité de la recherche en économie.

À cette fin, tous les paradigmes de la discipline doivent pouvoir se confronter sur le terrain scientifique, et cela sans intervention politique. Une fois ce constat établi, vous conviendrez que la notion d'orthodoxie a peu de sens. À cet égard, la recherche française en économie est dynamique, et cela est reconnu à l'échelle internationale. Je rappelle que Jean Tirole a reçu le prix de la Banque royale de Suède en mémoire d'Alfred Nobel en 2014, soit l'équivalent du prix Nobel en économie. Sur le fond, la recherche économique actuelle s'illustre en France et dans son cadre institutionnel actuel par une ouverture croissante à l'interdisciplinarité, notamment aux apports des sciences humaines et sociales. Ce qui est vrai des sciences humaines l'est également des sciences exactes, le lien entre l'économie, les sciences cognitives ou les mathématiques n'étant plus à prouver. Dans ces conditions, la création d'une nouvelle section, qui serait dédiée à l'économie « hétérodoxe » au sein du CNU ou du CNRS, n'aurait aucune plus-value. Il faut veiller à ce que le pluralisme devienne la règle, ce qui ne fera pas en séparant les tenants des différentes doctrines. Permettez-moi de rappeler également qu'il existe à l'heure actuelle plus d'une trentaine de sections du CNU dédiées aux sciences humaines et sociales. C'est également le cas au CNRS, qui comporte plusieurs sections. Là encore, il s'agit non pas de cristalliser telle ou telle théorie par rapport à telle autre, mais bien de garantir à chacun de pouvoir exercer son métier de scientifique, qui est de confronter les faits aux théories, afin de faire progresser la connaissance.

avis a été confirmé par Jean Tirole, qui a eu l'occasion de s'exprimer publiquement sur ce sujet. S'agissant de l'ouverture pluridisciplinaire du premier cycle universitaire en économie, cette filière bénéficiera comme les autres de la mise en oeuvre de l'enseignement modulaire et capitalisable dans les conditions prévues par la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, mais aussi par le projet du nouvel arrêté de licence en cours de rédaction.

dans une démarche d'économistes tout à fait respectables, mais qui relève de la pensée dominante en la matière. On a plus que jamais besoin, y compris pour notre démocratie, de pluralisme en matière de recherche et d'enseignement.

santé. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la situation tendue du groupe hospitalier du Havre, plus particulièrement de l'hôpital Pierre-Janet, qui en est l'hôpital psychiatrique. Depuis le 16 juin dernier, les agents de l'hôpital psychiatrique Pierre Janet sont en grève pour dénoncer l'absence de moyens suffisants pour prendre en charge les malades. Ce mouvement, initialement circonscrit aux urgences, s'est étendu à tout le pôle psychiatrie et santé mentale du groupe hospitalier. La situation critique dans laquelle se trouve l'établissement depuis plusieurs années conduit toutes les catégories de personnels soignants à tirer la sonnette d'alarme. En effet, le manque récurrent de personnel et l'absence d'investissements suffisants ne permettent plus d'accueillir les patients dans des conditions acceptables. Les urgences de nuit sont saturées, pour atteindre aujourd'hui un taux de 116 % de remplissage depuis plus d'une dizaine d'années. Depuis 2016, le plan Psychiatrie et santé mentale, doté de 15 millions d'euros pour les cinq prochaines années, prévoit la réhabilitation des trois pavillons : Boréal, Alizé et Caravelle. équivalents temps pleins ont été recrutés en 2017 et d'autres recrutements sont en cours. Malgré ces efforts, la situation demeure trop tendue et insuffisante pour que le service fonctionne normalement. De trop nombreux patients sont hospitalisés sur des matelas posés à même le sol, faute de lits en L'ARS a été sollicitée pour un accompagnement financier et des moyens matériels supplémentaires, sans réponse à ce jour. De plus, la demande de visite sur place de la directrice de l'ARS pour constater la situation est à l'heure actuelle toujours repoussée. Madame la ministre, comme à Saint-Étienne-du-Rouvray, les personnels au Havre sont à bout. Ils peuvent difficilement travailler et prendre soin des patients dans les conditions actuelles. À la veille de l'été, ils attendent des mesures concrètes, fermes et immédiates.

Comme de nombreux établissements de santé, le service d'accueil des urgences du groupe hospitalier du Havre connaît une augmentation croissante du nombre des passages aux urgences. La direction de l'établissement a décidé d'augmenter le personnel, avec un poste d'infirmier d'accueil et d'orientation. Par ailleurs, pour tenir compte des épisodes d'afflux saisonniers liés aux épidémies hivernales, l'agence régionale de santé accorde un financement spécifique depuis 2016 à l'établissement pour permettre des renforts temporaires durant la période hivernale, apport à hauteur de 500 000 euros en 2017. Parallèlement, l'agence régionale de santé travaille avec les représentants des médecins libéraux et les établissements pour renforcer la démographie médicale en Normandie, déploie dans ce cadre des pôles de santé libéraux et ambulatoires et s'engage dans la mise en oeuvre de communautés professionnelles territoriales de santé, qui ont notamment vocation à permettre d'améliorer la réponse aux demandes de soins non programmés en journée et, ainsi, de limiter l'impact sur les services d'urgence. Le groupe hospitalier du Havre a également engagé des coopérations renforcées avec l'offre de soins de ville au sein du SAMU, avec une expérimentation de régulation diurne portée par l'Association médicale des urgences havraises. Enfin, un nouveau cahier des charges de la permanence des soins ambulatoires sera adopté par la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie dans les prochaines semaines. semaines. Élaboré en concertation avec les professionnels et établissements de santé, ce cahier des charges renforcera les moyens médicaux consacrés à la régulation téléphonique. S'agissant de la psychiatrie, la direction de l'établissement a défini un plan d'action pour attirer et fidéliser des médecins psychiatres, repenser le rôle et la place des psychologues et des infirmiers, améliorer les conditions de travail des personnels et fluidifier les parcours des patients. Vous l'avez rappelé, le groupement hospitalier du Havre a aussi élaboré un ambitieux projet de restructuration immobilière des activités de psychiatrie. Toutes ces mesures visent à améliorer le fonctionnement Le groupement hospitalier du Havre est néanmoins confronté à un mouvement de grève engagé par les organisations syndicales depuis plusieurs semaines. Il est essentiel que le dialogue social reprenne au sein de l'établissement sur le fondement de toutes les améliorations que je viens de mentionner. La parole

de construire plus, plus vite et moins cher ; dans le même temps, les bailleurs sociaux disposeront de moins de moyens pour le faire. Surtout, les maires seront de plus en plus contraints par des prescriptions, notamment en matière environnementale, qui aboutissent à une raréfaction du foncier

dans cet hémicycle. Le premier amendement vise à limiter les règles de compatibilité entre les différents documents d'urbanisme aux seuls documents stratégiques des SCOT et des PLU, à savoir- excusez ces termes barbares ! -, pour le SCOT, le document d'orientation et d'objectifs, ou DOO,

possible de distinguer des zones de cohérence homogènes et, dès lors, de créer des plans de secteur permettant de mieux prendre en considération la diversité de nos territoires. Ces plans de secteurs définiraient les conditions d'aménagement de chaque zone, en garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères

Cette concordance pose un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, il faut que les PLUI soient compatibles avec les orientations du SCOT.

je souhaitais attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les difficultés rencontrées par l'association La Vie active et par l'organisme d'HLM Habitat Hauts-de-France dans la réalisation d'une résidence adaptée pour personnes handicapées dans la commune de Hersin-Coupigny, dans le Pas-de-Calais. Le terrain sur lequel doit se construire cette résidence se révèle être très pollué par les activités de son ancien propriétaire. Il s'agit d'un ancien site de la gare SNCF, racheté par la commune. Dans le cadre de cette vente, une étude de sols avait conclu à l'absence de pollution. Ce terrain a ensuite été vendu à la société Habitat Hauts-de-France, afin de construire quarante et un logements sociaux. À l'occasion du lancement des travaux, en avril 2015, cette société a découvert une trentaine de fûts contenant des hydrocarbures et enfouis dans le sol, le terrain étant lui-même très pollué. Habitat Hauts-de-France a procédé à l'évacuation d'une partie des fûts et à l'élimination des terres polluées, mais a fini par renoncer au chantier en raison du coût des travaux, qui atteignent déjà 600 000 euros. Face à cette situation, des réunions de concertation ont été organisées, regroupant l'ensemble des protagonistes. Malgré une proposition de prise en charge de la dépollution à hauteur de 50 % par le bailleur social, la SNCF refuse tout accord, ce qui bloque cet indispensable projet s'insérant parfaitement dans le cadre du contrat d'intérêt national du bassin minier.

que l'État a récemment missionné La Vie active pour la distribution de repas aux migrants. Monsieur le ministre, je souhaiterais connaître les initiatives que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour débloquer une situation qui n'a que trop duré.

La société Habitat-Picardie n'a pas souhaité donner suite à cette démarche, mais elle a indiqué à l'association qu'elle s'engageait à reprendre la construction des logements envisagés.

des rumeurs inquiétantes. Votre ministère aurait l'intention de supprimer 57 millions d'euros de crédits, dont 20 millions d'euros dès cette année. Vous le savez, ces centres répondent aux besoins les plus élevés en matière d'accompagnement. Les publics ayants droit sont ceux qui cumulent les détresses les plus fortes. Le temps de prise en charge est même jugé trop faible par de nombreux professionnels. Dès lors,

», votre projet de loi part du principe que ces familles pourront être locataires de logements privés ou publics avec un accompagnement modéré, nous n'obtiendrons plus de sorties positives. Tous les acteurs pourront vous le dire : le programme 177 souffre depuis bien trop longtemps d'une sous-budgétisation chronique. Chaque année, nous votons des crédits inférieurs aux enveloppes consommées durant l'année en cours.

l'aménagement du triangle de Gonesse, dont le projet Europa City constitue la première phase, répond à une attente forte des Valdoisiens et de leurs élus. Ce projet, développé par l'opérateur de l'État Grand Paris Aménagement, dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté constituée par arrêté du préfet du Val-d'Oise en 2016, est susceptible de créer 50 000 emplois et d'accélérer le développement économique de ce territoire, où sont situées trois des cinq communes les plus pauvres d'Île-de-France. Toutefois, l'avenir de ce projet est foncièrement lié à la desserte du site par la ligne 17 du métro automatique du Grand Paris. Cette ligne réduira le temps de trajet entre Roissy et Paris et desservira plusieurs territoires des trois départements qu'elle traversera. Elle permettra ainsi d'améliorer les conditions de mobilité des Valdoisiens et de faciliter leur accès à l'emploi. l'emploi. Or le Gouvernement semble vouloir retarder la construction de cette ligne. Certes, la loi de finances pour 2018 a définitivement acté le prêt de 1,7 milliard d'euros par l'État au consortium chargé de la construction de la liaison du Charles de Gaulle Express, laquelle est destinée aux touristes et aux voyageurs d'affaires, entre l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et la gare de l'Est. Mais cette ligne ne desservira pas les territoires qu'elle traversera. Pourtant, dans son discours de Bobigny, en 2016, le Président de la République déclarait : « La France des quartiers est aujourd'hui assignée à résidence, alors qu'elle veut réussir. Aujourd'hui, la facture du Grand Paris Express explose. Dès lors, certains axes semblent être remis à plus tard, notamment la ligne 17. Alors que la mise en service de la ligne était prévue dès 2024 jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle, et en 2030 jusqu'au Mesnil-Amelot, la nouvelle feuille de route du Grand Paris Express, dévoilée en février dernier, annonçait que les appels d'offres allaient être prochainement lancés pour vérifier la faisabilité technique d'une mise en service jusqu'au Bourget Aéroport à partir de 2024. La ligne ne devrait donc atteindre le triangle de Gonesse qu'en 2027 et l'aéroport Charles de Gaulle qu'en 2030 ! Monsieur le secrétaire d'État, quelle est votre position sur ce dossier ? Comment comptez-vous permettre au Val-d'Oise de disposer de toutes les clés nécessaires à son développement économique ?

Une partie de la ligne 17, que vous avez mentionnée, est concernée par ce rephasage. Ainsi, le Grand Paris Express arrivera en 2027 au triangle de Gonesse et en 2030 au Mesnil-Amelot. Le projet a donc pu être confirmé dans son intégralité, selon un échéancier désormais réaliste. Le budget consacré à la seule ligne 17 sera d'environ 40 millions d'euros en 2018 et de près de 900 millions d'euros d'ici à la fin du quinquennat. Tous ces éléments témoignent de l'engagement du Gouvernement pour la réalisation de cette infrastructure. Le Grand Paris Express accompagnera ainsi pleinement le projet d'aménagement du triangle de Gonesse, dont pourrait faire partie Europa City. Comme vous l'avez rappelé, le projet d'aménagement lui-même a pris un peu de retard. Le rephasage de l'arrivée de la ligne 17 au triangle de Gonesse ne nuira donc pas à la dynamique de développement de cette zone. En outre, une ligne de bus à haut niveau de service a récemment été créée entre la gare d'Arnouville, sur le RER D, et la gare du parc des expositions de Villepinte, sur le RER B. Elle dessert le site du triangle de Gonesse et offre ainsi aux Valdoisiens de nouvelles possibilités de déplacement, qui seront encore renforcées par la réalisation de la ligne 17. Enfin, il est important de ne pas opposer le Charles de Gaulle Express au Grand Paris Express, ou à tout autre projet de transports collectifs. Ces infrastructures répondent à des objectifs différents et sont donc parfaitement complémentaires. Certaines sont adaptées aux transports du quotidien, et donc financées sur fonds publics.

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vais vous parler, moi aussi, de l'enfermement que subit le département du Val-d'Oise, lequel est décidément bien mal loti en ce moment. Le 15 mai dernier, un mur de soutènement en terre armée de l'autoroute A15 s'effondrait sur le territoire d'Argenteuil. Il s'agissait d'un accident matériel, qui illustre le manque d'entretien du patrimoine autoroutier de l'État. L'effet de cet incident grave fut immédiat, compte tenu de la situation stratégique de cet ouvrage de l'A15, juste à l'entrée du viaduc de Gennevilliers dans le sens Cergy-Paris.

restent les seules ouvertes. Les premières études ont rendu leur verdict : aucun retour à la normale n'est attendu avant le début de l'année 2019. L'appel d'offres doit se dérouler cet été, et les travaux, qui

L'A15 et le viaduc de Gennevilliers sont un point de passage stratégique pour le sud et l'ouest de notre département. Face à l'extrême gravité de cette situation, qui s'installe dans la durée, un collectif d'élus, d'entreprises, et d'usagers s'est constitué le 27 juin dernier. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite savoir si l'État a bien pris conscience de l'impact économique et humain de cette situation sur notre territoire ; si l'État a bien prévu dans la procédure d'urgence de son appel d'offres que la réduction du délai des travaux constitue un critère déterminant dans le choix des entreprises et l'examen de variantes techniques, lesquelles peuvent avoir une forte influence sur la date de rétablissement de la circulation sur l'A15 ; enfin, si l'État est prêt à assurer la transparence sur ce dossier.

tout affaissement nouveau et sécuriser les interventions de réparation. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage aux agents du service public qui se sont investis sur ce chantier. Les travaux de réparation du remblai et de la chaussée commenceront dès la fin de l'été et devraient durer jusqu'au printemps de 2019.

anticiper cet accident ? Sachez que le patrimoine des ponts et murs du réseau routier national, non concédé en Île-de-France, est surveillé selon une méthodologie précise, comprenant la visite annuelle de chaque ouvrage et une inspection technique régulière, menée tous les trois ans. La dernière évaluation du mur de l'A15, en 2016, ne faisait apparaître aucun risque de dégradation et aucun défaut visible de stabilité nécessitant un entretien d'urgence. L'inspection détaillée périodique des éléments du mur était prévue pour 2019. Que compte faire le Gouvernement pour éviter de telles situations ? Le rapport du Comité d'orientation des infrastructures, infrastructures, remis en février dernier, insiste justement sur les priorités que constituent l'entretien et la régénération du réseau routier national non concédé ainsi que la modernisation de son fonctionnement. un terme à la dégradation du réseau, l'effort budgétaire consenti depuis 2015 doit être amplifié et stabilisé sur la durée. En 2018, un peu plus de 800 millions d'euros seront consacrés à l'entretien et à l'exploitation du réseau,

quantitatifs d'amélioration du réseau à échéances quinquennales en 2022, 2027, 2032 et 2037. Sachez en tout cas, en tant qu'ancien président du conseil départemental, que, sur ce dossier, le cabinet de la ministre des transports se tient à votre entière disposition, ainsi qu'à celle de l'ensemble des élus du Val-d'Oise.

Rosny-sous-Bois, commune de Grand Paris Grand Est, a avancé, la suite du parcours semble plus incertaine, alors que ce projet est acté par le décret n° 2011-1011 2011-1011 du 24 août 2011, qui approuve le schéma d'ensemble du nouveau réseau de transports en commun du Grand Paris. Si ce tronçon du Grand Paris Express ne voyait pas le jour, de nombreux projets immobiliers et zones d'activités pourraient en pâtir

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur Roger, permettez-moi d'excuser l'absence de la ministre des transports, qui m'a confié la charge de répondre à votre question. Le prolongement de la ligne 11 de Rosny-Bois-Perrier à Noisy Champs appartient au réseau complémentaire du Grand Paris Express. Il a été introduit dans le schéma d'ensemble établi par la Société du Grand Paris au titre des réseaux structurants. Il relève donc non pas de la maîtrise d'ouvrage de la Société du Grand Paris, mais de celle d'Île-de-France Mobilités. Le tracé de ce prolongement comporte une fourche à partir de Rosny-Bois-Perrier, avec une branche en direction de Champigny et une autre en direction de Noisy-Champs. Lors de la définition du schéma du nouveau Grand Paris, en mars 2013, l'option visant à réaliser cette seconde branche sous la forme d'un prolongement de la ligne 11 avait été envisagée, sous réserve d'études approfondies. Île-de-France Mobilités a donc confié à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme une mission en vue d'actualiser les données sociodémographiques prises en compte pour les études de ce prolongement, en lien avec les communes concernées. Ce travail a conduit à une légère amélioration des résultats, qui restent, malgré tout, négatifs d'un point de vue socio-économique. Face à des choix qui engagent des investissements publics importants, la démarche d'Île-de-France Mobilités, qui consiste à en évaluer la pertinence, apparaît légitime ; il lui revient de se prononcer sur leur opportunité.

Ce n'est pas une bonne méthode de travail avec les collectivités territoriales, qui, une fois de plus, sont méprisées. La

L'article 126 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique prévoit pourtant que, dans le cas d'investissements importants réalisés par les opérateurs industriels, les ouvrages ne peuvent être soumis à la concurrence. Or la Commission européenne conteste cette disposition et exige que la France renouvelle ses concessions hydrauliques, sous prétexte que la situation existante nuit à la concurrence auprès des clients finaux. Je rappelle que plus d'un million de nos concitoyens ont changé de fournisseur en 2017, preuve que la concurrence sur le marché de l'électricité existe déjà. Par ailleurs, les concessions hydroélectriques participent d'un service public d'intérêt général l'accès à l'électricité, qui est un bien de première nécessité pour tous nos concitoyens et qui doit donc rester une compétence exclusivement française. Cette ouverture à la concurrence menace également la gestion des multiples usages de l'eau, avec toutes les conséquences que cela peut avoir en termes environnementaux et sociaux, craintes quant aux autres spécificités et fonctions des barrages, telles que la sécurité, l'irrigation des cultures, l'alimentation en eau potable, la gestion des crues, l'approvisionnement des industries, que des inquiétudes sur le maintien des emplois directs et indirects locaux. Une telle décision risque, notamment, de compromettre le développement, voire la sécurité sanitaire, de la région Occitanie, déjà confrontée à un problème majeur de ressources en eau dans les années à venir.

pleinement de la transition énergétique. Le droit français, en conformité avec le droit européen, prévoit que les concessions hydroélectriques échues doivent être renouvelées par mise en concurrence. Cette situation est désormais ancienne, nous en héritons. La loi relative à la transition énergétique et ses textes d'application ont justement réformé le cadre du renouvellement des concessions électriques, en prévoyant la possibilité, pour les collectivités locales, d'être associées à la concession, notamment des sociétés d'économie mixte hydroélectriques, des SEMH. L'option de regrouper des concessions hydrauliquement liées pour faciliter leur exploitation et favoriser la sûreté répond à une demande des élus locaux, mais également du corps préfectoral pour la gestion des vallées. De nombreux échanges ont lieu avec la Commission européenne,

et de l'intérêt public. L'objectif est d'aboutir rapidement à une sortie du, qui nuit aux investissements dans le secteur pour chacun des ouvrages et constitue une source d'incertitude pour les entreprises, pour les salariés et pour les collectivités territoriales concernées. Le Gouvernement continuera donc à défendre les regroupements de concessions indispensables à la cohérence des vallées,

On s'y dérobe depuis des années, et il faut trancher ce problème, afin d'optimiser la gestion de nos barrages et de relancer l'investissement, tout en redistribuant des ressources financières vers les différents territoires. Le statut des personnels sera préservé dans tous les cas- il faut le dire encore, puisque des inquiétudes peuvent naître ici ou là -et les cahiers des charges devront prévoir la reprise des personnels par le nouvel exploitant, le cas échéant. Je rappelle enfin un fait intangible : les barrages appartiennent et continueront d'appartenir

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse, mais elle ne me satisfait pas tout à fait. Je rappelle que les grands barrages des Pyrénées, du Massif central et des Alpes sont à la base de notre politique énergie énergétique d'électrification, qu'ils font partie du patrimoine industriel national et qu'ils doivent donc rester français. En outre, vous l'avez dit, miser sur l'énergie hydraulique s'inscrit pleinement dans une perspective d'évolution vers les énergies renouvelables. EDF et les opérateurs historiques ont fait leurs preuves dans ce domaine. Pour ces deux raisons, il me semble important, en tant qu'élue de territoire, que les opérateurs historiques gardent la main sur notre production hydroélectrique, afin de préserver certaines garanties. Dans ma commune des Pyrénées, EDF gère deux barrages.

de santé publique ! Lors des multiples grèves du secteur hospitalier et médico-social, les hôpitaux psychiatriques ont dénoncé la dégradation de leurs conditions de travail et de l'accueil des patients, ainsi que le manque patent de moyens. La discipline connaît une paupérisation d'ampleur, alors même que les besoins ne cessent de croître. Entre 2010 et 2016, quelque 300 000 personnes supplémentaires ont en effet été suivies en psychiatrie ! Faut-il évoquer la nécessité de prévenir et de soigner

Les soins psychiatriques sont réduits à la prise en charge d'urgence, le recours à la chambre d'isolement s'accroît, conduisant la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté à évoquer « des pratiques indignes Le 26 janvier dernier, Mme la ministre a annoncé douze mesures en faveur de la psychiatrie. Si elle a indiqué ainsi la volonté du gouvernement de préserver les moyens, elle n'a pas évoqué d'augmentation des budgets dédiés,

sur lequel il faut évidemment agir le plus en amont possible. Cette question est certainement insuffisamment prise en compte dans notre pays jusqu'à présent, et la psychiatrie a été laissée à l'écart des différentes réformes. Le Gouvernement s'engage à changer de stratégie. La ministre des solidarités et de la santé a présenté, le 28 juin 2018, lors de l'installation du nouveau comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie, une feuille de route très ambitieuse, l'un de ses axes vise précisément à garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité. Pour organiser les parcours de soin des patients, chaque territoire devra se doter d'un projet territorial de santé mentale, auquel participeront tous les acteurs de l'organisation territoriale. Pour concrétiser ces ambitions, la ministre porte une attention particulière aux moyens de la psychiatrie, notamment de la pédopsychiatrie, qui est une discipline trop délaissée. Elle souhaite ainsi accroître le nombre de professionnels formés. Cela passe par les effectifs dévolus à la psychiatrie, mais aussi par le renforcement de la formation des médecins généralistes dans le champ de la santé mentale. Il faut promouvoir l'accès à des stages de formation en psychiatrie des étudiants en deuxième et troisième cycle. Par ailleurs, un travail sur les pratiques avancées en psychiatrie sera réalisé. Enfin, la ministre souhaite résolument développer la recherche dans cette spécialité. Afin que soient adaptées les ressources, une réflexion a été engagée début 2018 avec les agences régionales de santé pour concevoir des critères de modulation interrégionale. Celle-ci a déjà conduit à un renforcement de la dotation de trois régions historiquement sous-dotées. Parallèlement, des travaux sont menés sur la réforme des modes de financement. Il faut faire en sorte que les établissements de santé mentale soient incités à s'inscrire dans des démarches de qualité.

La médecine à l'école connaît une anémie profonde, qui conduit à une prise en charge inégale des élèves. En dix ans, le nombre de médecins scolaires a chuté de près d'un tiers. Si 57 % des enfants sont vus par un médecin pendant leur scolarité, l'amplitude des visites varie de 0 % à 90 % selon les départements. Vous-même, monsieur le ministre, avez reconnu, lors d'une audition au Sénat, que la visite médicale « n'était pas une réalité pour tous les élèves de France ». Nous sommes donc d'accord sur le constat.

parmi lesquelles Villeurbanne, Antibes, Bordeaux, Rennes, Grenoble, Vénissieux ou Lyon, qui disposent d'un service de médecine scolaire. Ceux-ci répondent aux besoins des enfants, qui sont parfois dans des situations de grande pauvreté.

et permettre, de ce fait, la réduction des inégalités sociales. Notre politique de santé repose sur trois axes : l'éducation à la santé, la prévention et la protection. Ces axes sont mis en oeuvre dans le cadre du parcours éducatif de santé, qui constitue un ensemble continu de la maternelle à la terminale, cohérent et progressif. Pour veiller à la santé des élèves et à leur bien-être, l'institution scolaire s'appuie sur les médecins et les infirmiers de l'éducation nationale, qui participent à la mise en oeuvre de ce parcours de santé, mais elle peut également recourir à d'autres intervenants. Le code de l'éducation, dans son article L. 141-1, lui fait obligation d'assurer à tous les élèves au cours de leur sixième et douzième année une visite médicale ou de dépistage, une prise en charge et un suivi adapté, notamment en prenant les mesures appropriées pour que les familles soient aussitôt informées des constatations médicales. Il est arrivé, en effet, que les collectivités prennent en charge cette mission pour l'école primaire, vous l'avez rappelé. Le ministère de l'éducation nationale leur verse alors une subvention. C'est encore le cas de onze villes, qui continuent à prendre en charge les missions de santé scolaire. Comme il s'agit d'une compétence de l'État, le versement de la subvention est assis sur une convention de délégation négociée par chaque service académique en tenant compte des spécificités locales. Or il n'est pas possible de comparer les dépenses des collectivités en la matière et celle de l'État, d'abord parce qu'elles ne concernent pas le même périmètre : les prestations des communes sont circonscrites au premier degré, tandis que celles de l'État concernent le premier et le second degré. De plus, et surtout, la plus grosse part de la dépense de santé scolaire du ministère de l'éducation nationale concerne les personnels c'est le salaire des infirmières, des médecins et des secrétaires médico-scolaires du premier degré comme du second degré. Toutefois, si certaines des communes déposaient des demandes argumentées réexamen des conditions de partenariat auprès des services rectoraux, ces dossiers seraient étudiés de manière approfondie ; à la suite de votre question, je vais examiner ce dossier avec attention. Bien entendu, cette évolution des rectorats se fera en liaison avec l'administration.

de langues étrangères à partir du CE1. À l'issue de cet enseignement, tous les élèves doivent avoir atteint le niveau 1 du cadre européen commun de référence des langues dans l'une des huit langues retenues. Pour chaque académie, dans le cadre de ses attributions, la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères veille, notamment, à la diversification de l'offre linguistique. Toutefois, force est de constater sur le terrain que de nombreux parents d'élèves s'émeuvent d'une situation réelle qui apparaît bien éloignée de la théorie. Dès 2011, j'avais interpellé le ministre de l'époque au sujet du manque de moyens accordés à la mise en place de l'apprentissage des langues au sein de l'école primaire. J'avais cité l'exemple d'une commune que je connais bien, celle de Talange, en Moselle, en évoquant le cas d'une école dans

Le directeur académique reconnaît par courrier que l'adéquation entre les besoins et l'offre est difficile à réaliser, compte tenu des contraintes techniques et financières auxquelles cette gestion est soumise. Pourtant, toutes les études s'accordent pour souligner que les premières années d'enseignement sont décisives dans l'apprentissage d'une langue. Si nous sommes conscients des difficultés réelles rencontrées par le monde enseignant en termes de moyens, la réponse du ministère de l'éducation nationale ne peut pas être satisfaisante : l'avenir de nos enfants ne saurait se trouver pris au piège des seules contingences matérielles ou financières

Dans le cadre d'un accord avec les autorités consulaires italiennes, l'enseignement de l'italien dans les deux écoles de la commune, ainsi qu'à Metz et à Moyeuvre-Grande, est assuré par trois locuteurs natifs, financés par le consulat. L'inspectrice de l'éducation nationale chargée de la circonscription du premier degré dont dépend Talange atteste la qualité de l'enseignement dispensé. L'apprentissage de l'italien permet d'élargir le répertoire linguistique des élèves et vise l'obtention du niveau A1 en italien en fin de CM2. L'inspectrice de l'éducation nationale chargée du dossier n'a fait part d'aucun retour négatif des familles au sujet de cet enseignement. Dans le cadre de la poursuite de la scolarité, la continuité linguistique est assurée au collège de Talange, qui offre dès la sixième une classe bilangue anglais-italien et l'enseignement de l'italien en langue vivante 2. La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères, présidée par le recteur de l'académie, est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, ainsi qu'à la cohérence et à la continuité des parcours. Cette commission établit chaque année un bilan de l'enseignement et peut proposer des aménagements à la carte académique des langues. Il est possible d'envisager,

je dois dire que les témoignages entendus à l'occasion de ma rencontre avec l'Association d'adultes et de parents d'enfants dyslexiques de l'Essonne semblaient en totale contradiction avec le discours officiel prononcé lors de la rentrée de septembre alors qu'avait été annoncé « le développement de l'information aux familles afin de simplifier leurs démarches », ces mêmes familles parlaient plutôt d'un parcours du combattant et de méandres administratifs. Alors que « le renforcement de l'accompagnement humain » avait été présenté comme une priorité, les familles faisaient état d'un handicap invisible et d'un manque de communication, parfois même de considération. D'ailleurs, la formation des enseignants sur les troubles spécifiques du langage et des apprentissages est primordiale. Enfin, alors que « le numérique au service d'une école inclusive » avait été vanté, ces parents dénonçaient une discrimination en constatant que leurs enfants se voyaient refuser pour des examens les aménagements auxquels ils étaient pourtant habitués en comme des ordinateurs, la présence d'auxiliaires de vie scolaire ou du temps supplémentaire. Certes, la scolarisation de ces jeunes aux besoins particuliers peut entraîner des difficultés pour l'administration ; je puis le concevoir. Toutefois, afin de les accompagner positivement dans leur parcours, il paraît légitime que des aménagements simples et pragmatiques soient mis en place pour simplifier la vie de ces nombreuses familles et soutenir ces enfants dans l'apprentissage des savoirs. Monsieur le ministre, cette situation m'en rappelle malheureusement une autre : celle, elle aussi souvent oubliée, des jeunes aidants. S'occupant chaque jour d'un parent malade ou handicapé, ils sont épuisés : ils ont donc besoin d'une meilleure adaptation et mériteraient de bénéficier également d'un accompagnement personnalisé. Cela devient urgent En conclusion, et sans remettre en cause la sincérité de vos propos ni votre engagement plein et entier, un décalage entre les souhaits et la réalité du quotidien est à déplorer. Or l'école de la République ne saurait négliger l'idéal d'égalité auquel nous croyons tous Pour reprendre les mots de Jacques Chirac, « la démocratie, c'est l'égalité des droits, mais la République, c'est l'égalité des chances ». Ainsi, la société inclusive qu'appelle de ses voeux le Président de la République ne peut s'affranchir d'une école qui soit elle aussi inclusive.

la priorité que constitue la réalisation de cette école inclusive. Depuis les propos tenus par Jacques Chirac voilà une vingtaine d'années, les choses ont beaucoup évolué, et dans un sens plutôt positif. Il faut considérer

C'est ce que l'institution scolaire s'engage à faire aujourd'hui et ce que nous avons pratiqué dans la période d'examen qui vient de s'achever. Dans l'intérêt même de l'élève, et afin de ne pas l'exposer à des conditions d'examen qui ne lui seraient pas familières, les aides et aménagements qui lui sont accordés doivent être en cohérence avec ceux qui lui ont été accordés tout au long de sa scolarité.